Face à ce phénomène, nous savons désormais que la stérilisation est la seule solution à la fois pérenne et efficace pour maîtriser les populations de chats, cette solution étant que par les associations de protection des animaux. Il va sans dire que les maires sont de plus en plus contraints de mettre en place des campagnes de stérilisation. Beaucoup d’entre eux indiquent se sentir seuls et démunis.

Toutefois, il est également autorisé de capturer, d’identifier, de stériliser, puis de relâcher les chats vivant en groupe. Cette solution présente l’avantage d’éviter la recolonisation des sites. Elle implique néanmoins un suivi de la population relâchée et suppose effectivement un budget pour la capture, les actes vétérinaires et l’alimentation des animaux. Son financement repose sur les mairies, avec l’appui éventuel d’associations de protection animale. C’est précisément le financement de ces opérations qui apparaît comme le premier frein à la mise en place du dispositif.

ont bénéficié de cette subvention. Le bilan des actions menées dans ce cadre sera effectué après l’échéance des conventions financières engagées avec les lauréats. Selon vous, madame la sénatrice, il resterait

largement utilisé en viticulture et en arboriculture pour la maîtrise des adventices. Malgré le renouvellement de l’autorisation de la flumioxazine par l’Union européenne jusqu’en 2037 et son autorisation continue dans d’autres pays européens, la France envisage d’interdire le Pledge dès 2025.

plaide unanimement pour le maintien de ce produit. Madame la ministre, allez vous aller contre la décision de l’Anses et aligner la position française sur celle de nos partenaires européens ? Par ailleurs, comment pensez vous résoudre l’impasse technique créée par cette interdiction, particulièrement dans les régions où l’alternative mécanique n’est pas viable ?

un seul produit de référence contenant cette substance, le Pledge, était autorisé pour désherber les vignes et les vergers. En décembre dernier, l’Anses a répondu défavorablement à la demande de renouvellement de l’autorisation de ce produit.

La Commission européenne, qui a été alertée sur ce sujet, n’a pas pris position. Ce n’est pas une issue satisfaisante. J’ai donc demandé à mes services d’identifier toutes les possibilités dont nous disposons pour renforcer l’harmonisation des autorisations.

Face à la raréfaction des solutions chimiques, je me suis impliquée, dès le jour de ma nomination, pour relancer les travaux du comité des solutions. L’objectif est d’identifier les produits dont peuvent bénéficier les producteurs des autres États membres et qui pourraient faire l’objet d’une autorisation en France. Ces travaux sont en cours et portent

Les défis climatiques ne pourront pas être relevés par un engagement partiel ou des initiatives trop isolées. Quels moyens comptez vous donner à cette mobilisation ? Comment entendez vous l’accélérer ?

la ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage pleinement votre préoccupation de faciliter l’émergence et la diffusion des solutions dans le cadre de projets de recherche expérimentale et déploie d’ores et déjà des actions d’une ampleur sans précédent. Dans le cadre du programme national de développement agricole et rural (PNDAR) 2022 2027, les programmes portés par les chambres d’agriculture,

Cette programmation constitue le cadre stratégique de développement et de massification que vous demandez, dont l’enseignement agricole est un partenaire incontournable. La stratégie Écophyto 2030,

Prise de risque amont aval et massification de pratiques visant à réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles » (Praam). Il vise à inciter au développement et à la mise en œuvre de systèmes de pratiques de protection des cultures reposant sur l’utilisation de combinatoires de leviers déjà éprouvés l’accompagnement de projets ciblant des acteurs économiques à l’échelle territoriale. En outre, des crédits alloués à la planification écologique ont également permis de renforcer le soutien de l’État aux innovations culturales et à leur massification.

Prenons l’exemple d’un projet immobilier de moins de 5 000 mètres carrés. Le premier paiement intervient 90 jours après l’achèvement des travaux, mais au sens fiscal, c’est à dire lorsque le propriétaire déclare le bien habitable, et non plus selon la logique urbanistique d’avant la réforme. Cette déclaration peut intervenir six ans après l’octroi du permis de construire. Si le montant de la taxe dépasse 1 500 euros, un second paiement intervient six mois plus tard, soit neuf mois après la fin des travaux.

Dans certains cas, il faut attendre jusqu’à six mois entre l’encaissement par l’État et le reversement aux communes. Résultat : des tensions de trésorerie, l’incapacité pour l’ordonnateur à établir un budget primitif sincère, faute de pouvoir anticiper les recettes, et une capacité d’investissement réduite dans des projets structurants. Avant la réforme, le calendrier était bien plus clair : 50 % de la taxe étaient appelés à douze mois et le solde était versé vingt quatre mois après l’autorisation d’urbanisme. Aujourd’hui, le nouveau système complique la gestion pour les collectivités, sans même garantir de meilleurs délais. Madame la ministre, d’autres solutions permettraient elles de mieux concilier les intérêts des collectivités locales et les impératifs de l’administration centrale ? Un calendrier clair est il envisageable ? Un retour à l’ancien système, plus lisible et prévisible pour les collectivités, serait il une option ? La simplification que nous recherchons tous ne doit pas se faire au détriment de l’efficacité globale. Les collectivités ont besoin de réponses précises, car, à ce rythme, elles risquent d’attendre le versement

le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la DGFiP s’est accompagné du report de la date d’exigibilité de celle ci. Cette date est dorénavant calée sur la réalisation définitive des travaux. Un système d’acompte a été créé, permettant de neutraliser les effets sur les ressources des collectivités, notamment pour les grands projets dont la construction s’étale sur plusieurs années. Le décalage de calendrier évite l’émission de taxes pour des projets abandonnés, qui induisaient auparavant une annulation de taxation et le reversement des sommes indûment perçues. Afin d’optimiser les délais, la liquidation de la taxe s’appuie sur la dématérialisation du processus déclaratif, la création d’un référentiel des délibérations des collectivités locales et l’automatisation du calcul des taxes d’urbanisme. Des dysfonctionnements opérationnels ont pu être observés à l’ouverture de ces services. La dématérialisation a en effet suscité des interrogations de la part des usagers et a abouti à des erreurs, ralentissant ainsi la liquidation des taxes. Afin d’éviter l’envoi de titres de paiement erronés, la DGFiP a mis en œuvre un système de vérification préalable, qui freine les envois et les paiements Un plan d’action pour améliorer la lisibilité du processus déclaratif a donc été élaboré et un parcours rénové est proposé depuis le 3 février dernier.

Rappelons cependant que les dépenses liées au transport sanitaire ont atteint 6,8 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 10,8 %, et qu’elles sont principalement financées par la sécurité sociale. Les taxis sont les premiers bénéficiaires de ces financements, représentant 41 % des dépenses de transports sanitaires en 2023, soit environ 2,8 milliards d’euros. À titre de comparaison, les ambulances en représentent 26 % et les véhicules sanitaires légers 13,5 %. À moyen et long termes, ces dépenses devraient continuer d’augmenter en raison du vieillissement de la population, de la hausse du nombre de patients atteints d’affections de longue durée bénéficiant d’une prise en charge à 100 à 100 % et du report du transport en véhicule sanitaire léger vers les taxis. Dans ce contexte, les discussions entre les organisations professionnelles et la Cnam doivent se poursuivre afin d’aboutir à un accord équilibré tenant compte des contraintes budgétaires actuelles et de la situation économique des artisans taxis.

Le Gouvernement reste attentif aux difficultés du secteur et poursuivra le dialogue avec les professionnels pour trouver des solutions adaptées aux défis actuels. La parole

Ce constat va à l’encontre d’un principe fondamental de l’Union européenne consistant à prioriser l’alimentation humaine et animale avant la valorisation énergétique. Par ailleurs, ce détournement fragilise le secteur, qui produit un excédent commercial de plus de 1 milliard d’euros, soit plus de 20 % du total de l’excédent commercial des entreprises françaises de l’agroalimentaire. Ce n’est pas rien dans un contexte économique très tendu. cette question légitime : pourquoi l’impact environnemental des graisses animales est il considéré comme nul dans le calcul de l’empreinte environnementale des biocarburants, alors qu’il est pris en compte pour les autres industries utilisant cette même matière première ? Le Gouvernement souhaite t il protéger l’utilisation de ces graisses dans les

La transition vers des énergies bas carbone est cruciale pour lutter contre le changement climatique et réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées. Les biocarburants jouent un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Pour limiter les éventuels conflits d’usage, en particulier en matière alimentaire, les réglementations française et européenne favorisent en particulier le développement des biocarburants avancés, issus notamment de résidus et de matières usagées. Je précise que les carburants fabriqués à partir des graisses animales de catégorie 3 ne sont pas considérés comme des biocarburants avancés et ne sont donc pas particulièrement favorisés. Ces graisses sont aujourd’hui valorisées dans différentes filières, dont celle de la nourriture animale, aussi bien pour les animaux de compagnie que le bétail.

Je vous confirme que la nourriture animale fait bien partie des usages prioritaires des graisses animales. Nous l’avons même inscrit dans l’ordre de mérite des usages de la biomasse. Cependant, le secteur de la nourriture animale ne saurait à lui seul valoriser l’ensemble de cette ressource. La valorisation en biocarburants représente une alternative pertinente permettant de valoriser les ressources non utilisées par l’alimentation animale.

la taxe foncière payée par les agriculteurs. Or les aménagements militaires étant exonérés de taxes, les ressources disparaissent entièrement. D’une façon générale, les communes ne tirent aucun bénéfice financier lié à la présence d’un terrain militaire.

je souhaite savoir quelles mesures de compensation pourraient être envisagées pour soutenir ces communes, non seulement dans ce cas précis, mais aussi pour d’autres territoires confrontés à des situations similaires ? La parole

Comme vous le savez, les bâtiments et terrains qui appartiennent à l’État sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties lorsqu’ils sont affectés à un service public, ou sont d’utilité générale, et ne produisent aucun revenu. Ces conditions sont cumulatives et s’apprécient à l’égard du propriétaire, en l’occurrence l’État. Sur ce fondement, les terrains ou bâtiments, les champs de manœuvre et les casernements utilisés par les armées pour le service public de la défense nationale sont exonérés de la taxe foncière. Néanmoins, la présence sur le ressort géographique communal d’immeubles affectés à un service public ou d’utilité générale crée des externalités positives, notamment des retombées fiscales indirectes. Ainsi, la présence de logements accueillant des familles de militaires vient renforcer la population et donc l’activité économique. des milliers de militaires et des dizaines de civils, la base militaire aérienne de Bricy constitue un vivier d’emploi et une source d’activité économique importante pour les communes alentour. J’en viens à l’extension des bases aériennes sur des terres agricoles. Dès lors qu’ils font l’objet d’une amodiation autorisant par exemple la récolte des herbes ou le pacage des animaux, les terrains militaires sont considérés comme productifs de revenus et sont donc assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

70 millions d’euros d’investissement sur cinq ans, ainsi que des volumes de production minimaux pour les produits sensibles, notamment le Doliprane, sont également prévus. Nous avons souhaité et obtenu l’entrée de Bpifrance au capital d’Opella afin de disposer d’un droit de regard sur la stratégie de l’entreprise et d’y faire valoir nos intérêts, au service de notre souveraineté.

par le biais de l’authentification numérique, elle a toutefois reporté sur les utilisateurs une contrainte de possession et de bonne utilisation des téléphones portables. Bien que les dispositions de l’article L. 311 9 du code monétaire et financier prévoient notamment que « le client peut, immédiatement et à n’importe quel moment de la relation contractuelle, s’opposer par tout moyen à l’usage

le téléphone portable pour accéder à son compte en banque crée une fracture numérique. Cette obligation, qui diffère drastiquement d’une banque à l’autre selon les services clients, pèse notamment sur les personnes âgées ou fragilisées, qui ne possèdent pas de téléphone et ne sont pas formées à

Je vous remercie

de ces tarifs réglementés. Dans un contexte de forte hausse du coût de l’énergie, les tarifs réglementés de vente d’électricité, plus protecteurs que les tarifs libres, sont essentiels pour protéger les petites entreprises, les collectivités locales et les particuliers. À défaut, ceux ci peineraient à poursuivre leur activité ou à boucler leur budget.

a affirmé son soutien au dispositif Territoires d’industrie et sa volonté de reconduire le dispositif Rebond industriel. Je souhaite insister sur les besoins de financement

dans la stratégie industrielle de la France. Lancé en 2018 et confirmé dans sa phase 2 en 2023 par le Président de la République, ce dispositif cofinance notamment un réseau de chefs de projet chargé d’animer la gouvernance des projets en lien avec les élus et les industriels.

décroissent, le nombre de demandes de logements augmente, les programmes urbains sont en forte expansion et l’augmentation des inscriptions en crèche ou dans les écoles est parfaitement tangible.

le recensement est mené en partenariat entre l’Insee et les communes. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, la population est calculée par l’Insee uniquement à partir des informations recueillies par les communes : le nombre de logements issu du répertoire d’immeubles localisés et le nombre moyen de personnes par logement issu des enquêtes effectuées auprès des habitants. Les communes sont donc à l’origine des informations utilisées pour le calcul des populations. Les nouvelles constructions sont par exemple bien prises en compte dans le répertoire susvisé, qui est mis à jour en continu à partir des permis de construire et que les communes peuvent amender à tout moment.

de référence. Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les communes, qui ne sont pas recensées la même année, la population publiée à la fin d’une année reflète actuellement la situation au milieu du cycle quinquennal de recensement, soit la situation effective

la Cnerp vient d’approuver la réduction de ce décalage à deux ans, délai qui a été reconnu comme le meilleur équilibre entre « fraîcheur » et robustesse des données.

grâce à l’exploitation de leurs ressources, la Guyane française demeure dans un état de précarité et de pauvreté, non par manque de richesses, car elle dispose des mêmes ressources que ses voisins, mais parce que des décisions centralisées entravent toute dynamique de développement, maintenant la Guyane sous cloche. La Guyane est en effet asphyxiée par des réglementations excessives et inadaptées, un accès au foncier verrouillé et des projets bloqués au nom d’une protection environnementale, qui, paradoxalement, favorise l’exploitation illégale et l’économie souterraine, qui n’ont que faire des critères écologiques. résultat une population privée d’emploi et de perspectives, un sentiment croissant d’injustice, incitant même à la révolte. Comment en effet expliquer à la population guyanaise que son territoire souffre d’une économie moribonde, alors que celui ci est riche de ressources au grand potentiel économique ?

Ne pensez vous pas qu’il est temps de reconsidérer la position de l’État pour assurer le développement durable de la Guyane, dans le respect de ses écosystèmes, cela va sans dire, mais aussi de ses propres besoins de plus en plus pressants ?

notamment pour permettre l’orpaillage légal. En matière de simplification des normes, notre pays dispose d’importantes marges de progression. Le projet de loi de simplification de la vie économique adopté en première lecture par le Sénat

Malgré le recrutement de plus de 4 000 accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) depuis 2017, trop d’élèves se retrouvent sans solution, tandis que d’autres élèves sont insuffisamment accompagnés dans un milieu qui n’est pas adapté à leurs besoins, ce qui les expose à des situations de détresse pouvant engendrer de la violence contre eux mêmes ou contre leurs camarades, comme cela s’est produit à l’école élémentaire Les Halbrans, à Pont Saint Martin, en Loire Atlantique. En 2023, le gouvernement d’alors a lancé un acte II de l’école inclusive, incluant la revalorisation du métier d’accompagnant, l’augmentation

Ces équipes interviennent en prévention et le plus en amont possible d’un risque de rupture de parcours. Tout est donc mis en œuvre pour permettre un accompagnement plus fluide, des réponses plus rapides et une meilleure articulation entre l’éducation nationale et le secteur médico social. Cette année, nous irons plus loin en créant plus d’une centaine de nouveaux pôles d’appui à la scolarité sur tout le territoire. Chaque famille doit en effet pouvoir compter sur un accompagnement efficace,

– il faut avoir obtenu une note supérieure à dix pour pouvoir valider la sixième année d’études –, mais aussi classante. Force est de constater que les modalités de ce concours national renforcent les déserts médicaux sur notre territoire. En 2024, lors des épreuves de l’Ecos, plusieurs dysfonctionnements ont été révélés

Dans d’autres pays, cet oral est validant, il n’est pas validant et classant. Je vous demande donc, monsieur le ministre, si vous envisagez de rendre cet examen uniquement validant, plutôt que validant et classant.

nous avons urgemment besoin de médecins. Plusieurs candidats auraient été arbitrairement recalés en raison d’une suppression injustifiée de postes par le jury. Alors que nous appelons tous à la régularisation des Padhue, indispensables au fonctionnement de nos services de santé, l’administration joue une partition inverse et pour le moins curieuse. Qu’en est il, monsieur le ministre monsieur le ministre de médecine en 2024. Elle a été construite en concertation avec les associations de représentants d’étudiants, en particulier. Son objectif était de permettre une évaluation non seulement sur des connaissances, mais aussi sur des compétences. Le nouveau concours met ainsi en place des épreuves dématérialisées nationales, dites EDN, réalisées sur tablette, et des examens cliniques objectifs structurés, dits Ecos. Les Ecos évaluent la capacité des étudiants à agir en milieu professionnel à travers leur savoir faire et leur savoir être, évidemment essentielles pour de futurs médecins. Les évaluations sont réalisées par deux examinateurs et sont standardisées grâce à une grille très précise limitant, autant que faire se peut, les risques de subjectivité.

des ajustements ont pu être apportés pour les épreuves réelles, qui se sont déroulées sans difficulté du 28 mai au 29 mai 2024, simultanément pour 8 000 étudiants dans trente deux facultés de médecine. Aujourd’hui, il n’y a pas de raison de remettre en question le caractère classant de cette épreuve clinique, car elle évalue des compétences différentes et complémentaires de celles des épreuves écrites. Par ailleurs, le caractère national des épreuves est indispensable pour garantir un classement équitable des étudiants à partir d’épreuves identiques. À l’issue de ce concours, une répartition par région et par spécialité est réalisée, qui tient notamment compte de la démographie médicale et des besoins en santé des territoires que vous avez très justement soulignés,

demeure la priorité du pays. J’en veux pour preuve l’annulation de la suppression de 4 000 postes d’enseignants. C’est un choix politique assumé, malgré le contexte budgétaire et la baisse du nombre d’élèves.

soit environ 1,6 % des effectifs, avec pour conséquence directe des classes un peu moins chargées. Ainsi, en 2017, une classe seine et marnaise comptait en moyenne 24,2 élèves contre 23,1

en situation de handicap durant le temps de pause méridienne. En effet, malgré son adoption à l’unanimité, la mise en œuvre de la loi a été entravée,

dans des conditions sur lesquelles nous pourrons revenir. L’ancienne ministre de l’éducation nationale, Mme Anne Genetet, a annoncé le 2 décembre dernier la publication prochaine d’un décret visant à simplifier la procédure administrative instaurée par la note de service du 24 juillet.

Chaque situation est étudiée en s’appuyant sur les recommandations des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ainsi que sur l’expertise des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial) et des pôles d’appui à la scolarité (PAS). Les familles sont associées à l’organisation de la temporalité de prise en charge de l’enfant. La seconde priorité, c’est de simplifier et de sécuriser le dispositif. C’est pourquoi un décret a été présenté au comité social d’administration du ministère de l’éducation nationale (Csamen), le 21 janvier dernier, afin de clarifier les règles et de faciliter la mise en place de cet accompagnement sur la pause méridienne. L’État assumera pleinement ses obligations en tant qu’employeur, garantissant ainsi aux familles, lorsque cela est jugé nécessaire, une prise en charge stable et efficace. Monsieur le sénateur, notre ambition est claire – et je crois qu’elle est partagée – : permettre à chaque élève en situation de handicap d’avoir un accompagnement adapté à ses besoins et à son degré d’autonomie, tout au long de la journée. La parole

Malgré quelques assouplissements, notamment pour les réservistes de l’armée, il y a eu en réalité peu d’évolutions concrètes. Aujourd’hui, ces restrictions apparaissent dépassées au regard des progrès de la médecine. En effet, il est désormais possible de surveiller sa glycémie grâce à des lecteurs qui permettent de prévenir un déséquilibre. Les risques sont alors beaucoup mieux maîtrisés. l’état de santé prévoit la mise en place d’un comité interministériel d’évaluation. Les décrets nécessaires pour former sa composition ont été pris très tardivement. Ce comité doit, ou plutôt devait, rendre un rapport au Gouvernement et au Parlement tous les ans.

et porte sur un enjeu de justice sociale et d’égalité des chances. Comme vous l’avez rappelé, la loi du 6 décembre 2021 a institué un comité d’évaluation des textes encadrant le marché du travail. La composition de ce comité a été fixée par le décret du 22 avril 2022 et finalisée par l’arrêté du du 29 juin 2022, de manière à pouvoir évaluer la réglementation en vigueur et à en apprécier la pertinence à la lumière des avancées médicales et scientifiques afin de formuler des propositions.

Ces rapports permettent d’apprécier les avancées qui sont réalisées dans l’évaluation des conditions d’accès à certains métiers comme ceux des corps actifs, notamment de la police nationale. L’évolution des connaissances sur le diabète et les progrès technologiques pour améliorer les moyens de surveillance

ans plus tard, aucun gouvernement n’ayant agi vraiment, ni même vraiment agi, et ce malgré nos interpellations régulières, la situation n’a fait qu’empirer. et des statistiques (Drees), un service de votre ministère, montre que le desserrement du ne réglera en rien les problématiques de disparité de répartition des médecins sur le territoire. Cette même étude confirme que la situation ne sera réglée ni en 2030, ni en 2040, ni en 2050. On ne peut donc qu’espérer que des mesures fortes soient enfin prises, un jour, par un gouvernement et que soit mise en place une régulation à l’installation des médecins pour apporter des solutions concrètes à cette problématique. Rappelons que de telles mesures ont produit leur efficacité dans d’autres pays où elles ont été expérimentées, et même en France pour des professions de santé autres que les médecins. Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement envisage enfin de changer de braquet et d’agir vraiment en prenant les mesures qui s’imposent pour résorber les inégalités territoriales en matière d’accès aux soins.

aux soins. Monsieur le ministre, les chauffeurs de taxi conventionnés sont très mobilisés contre le projet de réforme de la convention cadre qui a vocation à s’appliquer pour les cinq prochaines années entre la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et les organisations syndicales représentatives.

la convention impose des conditions plus strictes pour ce qui est des tarifs et des critères de qualité de service. Le texte envisage en effet une tarification prévue à la baisse, une obligation de pratiquer le taxi partagé, ainsi que celle de respecter le trajet le moins onéreux possible, avec l’état de santé du malade. Les taxis dans nos territoires vivent essentiellement du transport professionnalisé, qui représente une part très significative de leur chiffre d’affaires.

comment le Gouvernement entend il prendre en compte la situation particulière des taxis qui ont une activité de transport sanitaire, notamment ceux qui travaillent en milieu peu dense ? La parole est à M. le ministre.

à l’avenir de notre système de santé. Pour que les jeunes médecins soient de plus en plus nombreux à choisir cette voie et à s’installer dans nos territoires, en 2022, une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale Cette période de consolidation doit notamment faciliter et sécuriser l’installation des jeunes médecins, en particulier dans les zones les moins dotées en professionnels de santé. Vous le savez, cette mesure est attendue avec impatience. Pourtant, les décrets d’application dont la publication était initialement annoncée pour juin 2023 n’ont toujours pas été publiés. Le 15 mai 2024, à l’occasion d’une séance de questions orales, ici même, le ministre Valletoux avait pourtant assuré une publication d’ici à la fin de l’été 2024. Alors que cette quatrième année doit entrer en vigueur dans le courant de l’année 2026, il est urgent de publier ces textes réglementaires. Leur absence freine la préparation des médecins généralistes encadrants, des futurs docteurs juniors, mais aussi celle des collectivités territoriales, qui doivent anticiper des enjeux majeurs tels que la rémunération, l’accueil, les lieux de consultation ou encore les logements.

pour la réplique. Monsieur le ministre, je ne doute absolument pas de votre engagement sur le sujet. Je vous entendais dire ce matin sur une chaîne d’information qu’il fallait rétablir la confiance.

de l’accès aux soins. Monsieur le ministre, tous les mois, nous découvrons avec effroi qu’un nouveau centre de santé risque de fermer. Ainsi, le Conseil de Paris débat cette semaine de l’avenir des centres de santé Réaumur, Stalingrad et de l’Institut mutualiste Montsouris. La situation critique de ces trois établissements fait écho à ma question sur les centres de la Croix Rouge française en Île de France. Ces centres, qui prennent en charge plus de 40 000 patients sans dépassement d’honoraires, ont fermé au mois de mai dernier après cessation de paiements. Les maires concernés, les élus de Paris et les organisations syndicales se sont exprimés contre la cessation de ces centres à un acteur privé à but lucratif

Ainsi, ces risques de fermeture mettent en lumière l’insoutenabilité du modèle actuel des centres de santé, notamment pour financer les missions à destination des plus vulnérables, c’est à dire celles et ceux qui nécessitent davantage de soins.,

Dans la Nièvre, le système hospitalier – en particulier les services d’urgence – traverse depuis des mois des difficultés majeures, qui compromettent gravement la prise en charge des patients, mettant leur vie en danger. Les exemples de défaillances sont nombreux et se répètent sans cesse, mois après mois, année après année. Celles ci donnent lieu à des situations de plus en plus dramatiques, dont certaines ont malheureusement conduit des Nivernais

vitale, aurait dû être rapide, ce patient s’est heurté à un enchaînement de défaillances. Il ne doit son salut qu’à la ténacité de sa famille, qui lui a fait parcourir 70 kilomètres, soit plus d’une heure de route, pour atteindre l’hôpital de Moulins. Là, il a enfin été diagnostiqué d’un AVC, mais trop tard pour bénéficier d’un traitement thrombolytique.

Nivernais et Nivernaises. Quelles mesures le Gouvernement envisage t il pour améliorer l’accès aux soins d’urgence dans la Nièvre, en particulier dans les établissements hospitaliers de Cosne Cours sur Loire, de Nevers, de Decize et de Clamecy et pour garantir que chaque patient bénéficie d’une prise en charge adaptée, rapide et sécurisante ?

estimait que faire une chose de la même manière et s’attendre à un autre résultat était une forme de lâcheté. Mes chers collègues, ne soyons pas lâches ! Il est temps de ne plus fermer les yeux sur la répétition incessante des mêmes erreurs. Nous devons agir sans délai pour apporter des changements concrets et garantir à chaque Nivernais un accès aux soins qui respecte sa dignité et sa vie.

durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Si ce dispositif a constitué une avancée majeure en facilitant l’accès à des psychologues conventionnés, plusieurs limites persistent : un financement insuffisant, une accessibilité inégale selon les territoires et des délais d’attente trop longs. Ces obstacles entravent une prise en charge rapide et efficace des personnes en détresse. La pandémie de covid 19 a laissé des séquelles profondes sur la santé mentale de notre population, plus particulièrement chez les jeunes. L’isolement, les perturbations scolaires et les incertitudes professionnelles ont entraîné une augmentation préoccupante des troubles anxieux, dépressifs et comportementaux. Ainsi, de nombreuses études soulignent que les besoins en accompagnement psychologique n’ont jamais été aussi élevés. les jeunes rencontrent encore de nombreuses difficultés pour bénéficier d’un suivi adapté. Le nombre insuffisant de professionnels disponibles et l’absence de structures adaptées dans certains territoires constituent des freins majeurs. Il est donc impératif d’augmenter les moyens alloués au dispositif, de revaloriser le tarif des consultations et d’améliorer le maillage territorial des professionnels de la santé mentale. L’adolescence et le début de l’âge adulte sont des périodes charnières, marquées par des transitions scolaires, sociales et professionnelles qui peuvent être source de stress et d’angoisse. Un suivi psychologique accessible et adapté est donc indispensable pour prévenir les situations de détresse conduisant à l’échec scolaire, à l’isolement ou, dans les cas les plus graves, à des conduites à risque. Au surplus, la question du bien être mental des jeunes ne peut être dissociée des défis sociaux auxquels ils sont confrontés : précarité économique, pression scolaire, manque de perspectives professionnelles…

je vous remercie de cette question extrêmement précise sur le régime indemnitaire des directeurs par intérim d’établissements d’hébergement pour personnes âgées

prime de fonctions et de résultats, lorsque l’intérim est assuré dans un autre établissement. Ces situations d’intérim sont malheureusement en hausse. On dénombrait 1 591 directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico sociaux en activité au 1 janvier 2023, contre 1 865 en 2013, soit une

Comme vous le savez, le complément de traitement indiciaire (CTI) issu des accords du Ségur de la santé de 2020 est une mesure de revalorisation salariale ayant vocation à reconnaître l’engagement, le dévouement et l’utilité sociale de l’ensemble des professionnels des établissements et services sociaux et médico sociaux Il leur donne droit à une prime de 189 euros net mensuels. Initialement réservée aux seuls agents des hôpitaux et Ehpad, la prime dite Ségur a été progressivement étendue et rendue obligatoire à d’autres structures et personnels. À date, l’ensemble des catégories d’agents publics y sont éligibles au sein des centres hospitaliers et des Ehpad, ainsi qu’une majorité des personnels des établissements et services sociaux et médico sociaux publics autonomes. Toutefois, au sein de ces derniers, une exception subsiste

Cette inégalité de traitement crée une disparité injustifiée entre personnels selon leur établissement d’affectation, qui concernerait entre 2 000 et 5 000 agents.

tous les professionnels du secteur social et médico social public autonome ? La parole

Toutefois, cette disposition n’a pas été retenue pour les personnels administratifs et techniques des ESSMS autonomes de la fonction publique hospitalière, qui sont principalement rattachés à des établissements publics départementaux Il s’agissait de garantir l’unicité des statuts des personnels relevant d’un même établissement hospitalier, tout en tenant compte des spécificités des métiers selon qu’ils s’exercent en milieu hospitalier ou sous l’autorité d’une collectivité territoriale.

la proposition de loi, le Gouvernement a présenté et fait adopter un amendement tendant à préciser que « les conditions et modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret,

d’autre part, restreindre le financement du permis moto le CPF compromettrait les professionnels de nombreux secteurs pour lesquels la mobilité est essentielle, notamment la livraison, les soins à domicile et divers métiers commerciaux. Les organisations professionnelles représentant les services de l’automobile

par an pour les travailleurs peu ou pas qualifiés. Le CPF est un levier essentiel pour acquérir des compétences nouvelles. Tous les permis sont éligibles au CPF depuis la loi du 21 juin 2023 qui en porte application. Les partenaires sociaux ont été dûment consultés en amont de l’encadrement. La Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) s’est d’ailleurs tenue le 17 avril 2024.

Durant les six premiers mois de 2024, les permis moto A1 ont représenté moins de 3 % des permis moto financés par les droits CPF des titulaires. La quasi totalité des permis moto financés le CPF concernent des motos de grosses cylindrées – jusqu’à 35 –, par exemple les Harley Davidson. En outre, les permis poids lourd et remorque restent éligibles au CPF et finançables avec les droits des titulaires. La parole est à Mme Annick Billon,

à la défense de la filière pêche ? Quelles actions entend il mener pour s’opposer à de nouvelles fermetures du golfe de Gascogne ? La parole

en 2023 à 273 en 2024, malgré le mois sans pêche. C’est là la démonstration éclatante que la pêche n’est pas la principale responsable des échouages. des échouages. Il est contesté, ensuite, pour des raisons écologiques. Alors qu’elle importe déjà 80 % de sa consommation de produits aquatiques, la France sera encore un peu plus dépendante des importations avec des produits de provenances toujours plus lointaines. C’est une aberration écologique. contesté, enfin, pour des raisons économiques. En effet, le mois sans pêche prive des milliers de mareyeurs, de transporteurs et de poissonniers du fruit de leur travail, tandis que la seule indemnisation de l’État ne permet pas de compenser leurs lourdes pertes. Cela fragilise grandement l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et menace la pérennité des emplois de toute Madame la ministre, ma question est très simple : comment le Gouvernement compte t il mettre un terme à ce dispositif du mois sans pêche, qui risque d’anéantir la pêche française sans pour autant sauver les dauphins du golfe de Gascogne ?

Le Gouvernement envisage t il de revoir le projet de révision du barème de MaPrimeRénov’ concernant ce type de chauffage ? La parole est à Mme la ministre.

installations de chauffage au bois domestique à haute efficacité énergétique. Elles doivent permettre de remplacer les équipements les moins performants et les plus polluants tels que les chaudières au fioul, mais également le chauffage au bois en foyer ouvert, inefficace, dont le rendement est

toujours possible de percevoir une aide de 4 000 euros pour l’acquisition d’une chaudière biomasse en remplacement d’un chauffage carboné. En 2025, les ménages les plus modestes pourront ainsi bénéficier d’un soutien

à nos consulats rappelant notamment que la présentation d’un titre valide ou périmé depuis moins de cinq ans et ne présentant aucun signe manifeste qu’il ait été délivré par erreur suffit pour prouver la nationalité française du demandeur et ne pas exiger de CNF, quel que soit l’acte demandé. De toute évidence, cela n’a pas résolu le problème, puisque la présentation d’un CNF est toujours exigée dans le cadre de simples démarches administratives comme le renouvellement d’un titre d’identité, de voyage, ou la transcription d’un acte d’état civil. civil. De nombreux usagers, qui possèdent pourtant la pleine et entière nationalité française, se lancent alors dans une démarche longue et complexe auprès du tribunal judiciaire pour obtenir cette preuve de nationalité. Beaucoup se heurtent à un refus pour des motifs purement formels comme l’oubli de joindre un document de cocher une case. D’ailleurs, les statistiques du ministère de la justice montrent que le taux de refus est passé de 69 % à 80 % entre 2018 et 2023. Dans plusieurs circonscriptions consulaires, nous observons qu’un refus de CNF peut avoir des conséquences dramatiques telles que la radiation du registre et de la liste électorale, ou, pis encore, le retrait d’un titre d’identité ou de voyage. Je pense à cette mère de famille en Inde, française par filiation, dont le renouvellement du passeport a été refusé en raison d’un refus de CNF et qui risque, avec toute sa famille, de se retrouver en situation irrégulière dans son pays de résidence, l’Inde ne reconnaissant pas la double nationalité. Ce n’est malheureusement pas un cas isolé. et des affaires étrangères ne dispose d’aucune donnée chiffrée sur le nombre de CNF sollicités par les postes consulaires. Ne serait il pas temps de mettre en place un indicateur lui permettant d’avoir une vision globale des pratiques dans nos consulats, de manière à éviter que certains ne procèdent à une demande systématique de CNF, suscitant le désarroi d’usagers dont la qualité

à l’ensemble du réseau des ambassades et des consulats. Cette note distingue les usagers titulaires d’éléments de possession d’état de Français consolidée et ceux qui ne peuvent en justifier.

Certes, depuis 2017, la procédure d’évacuation forcée permet aux préfets, saisis en ce sens et dans un délai de quarante huit heures après le dépôt de plainte, de mettre en demeure les squatteurs de quitter le logement.

Ce texte est donc perfectible, ne serait ce que parce qu’il ne dissuade absolument pas les squatteurs. Les violations de domicile sont toujours aussi nombreuses et les travaux de remise en état toujours aussi onéreux pour les victimes de cette infraction, qui sont donc doublement pénalisées. Aussi, afin que cet arsenal juridique soit davantage dissuasif, n’est il pas temps d’envisager une plus grande sévérité dans les peines encourues ainsi que de lourdes sanctions financières pour tout contrevenant à la loi sur la propriété privée ?

Par ailleurs, le législateur a créé aux articles 315 1 et 315 2 du code pénal deux nouveaux délits protégeant la propriété immobilière : d’une part, l’introduction ou le maintien illicites « dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel part, « le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d’habitation en violation d’une décision de justice ». En outre, les quanta des peines encourues du chef de sous location illicite ont été augmentés et un nouveau délit de propagande en faveur de ces comportements a été créé à l’article 226 4 2 1 du code pénal. Dans le prolongement de cette loi, le garde des sceaux a invité, dans une circulaire datée du 23 novembre 2023, les procureurs de la République à mettre en œuvre une politique pénale empreinte de fermeté.

La loi du 27 juillet 2023 a étendu cette procédure au squat de tout local à usage d’habitation, alors que, auparavant, seul le squat d’un domicile était concerné. Par ailleurs, les démarches administratives pour la personne concernée et le constat de l’occupation illicite ont été simplifiées.

Dans le cadre de la justice de proximité, ce tribunal a pu bénéficier de renforts significatifs en recrutant au fil de l’eau sept contractuels de catégorie A de 2021 à 2024, cinq juristes assistants et deux chargés de mission. Cela a permis d’améliorer la situation, qui demeure toutefois tendue. C’est pourquoi les effets des annonces du 28 mars dernier sont désormais très attendus. Ce jour là, à Annecy, Éric Dupond Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice, a concrétisé la dernière phase des recrutements de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, dite LOPJ, en dévoilant la répartition des effectifs supplémentaires au sein de toutes les juridictions. Le tribunal judiciaire de Tarascon pourra compter sur deux postes de magistrat du siège, deux autres au parquet, deux postes de greffier, deux postes de contractuel de catégorie A, attachés de justice. Ces créations sont indispensables pour renforcer cette juridiction, qui doit se montrer à la hauteur des missions qui lui sont assignées et répondre aux fortes attentes de nos concitoyens. Il importe à la fois de pérenniser les postes créés et de voir aboutir ceux qui ont été annoncés. Monsieur le ministre, pouvez vous me confirmer le maintien de la trajectoire budgétaire de recrutement ? Pouvez vous également me préciser le rythme de mise en œuvre ? Le tribunal de Tarascon peut il espérer de nouveaux postes en 2025 ? La parole est

avec les quatre créations de poste prévues entre 2023 et 2025. Enfin, s’agissant des effectifs de greffe, l’effectif cible du tribunal judiciaire de Tarascon est fixé à cinquante quatre agents à ce jour, dont vingt huit greffiers, auxquels s’ajouteront deux nouveaux greffiers à l’horizon 2027. Au 1 février 2025, un poste de directeur des services de greffe judiciaires, un poste d’adjoint administratif, un poste d’adjoint technique et un poste de contractuel B recruté dans le cadre de la justice de proximité demeurent vacants.

Voilà donc de nouveaux motifs de satisfaction, je vous en remercie, monsieur le ministre. Le tribunal de Tarascon pourra ainsi rendre une justice plus sereine.

à des conditions assez simples, de fabriquer puis d’assembler une arme fantôme. L’imprimante est capable de créer, grâce à des plans disponibles gratuitement et facilement sur internet, des pièces en plastique comme la crosse,

Il nous semble donc indispensable de mettre en place des mesures urgentes permettant d’endiguer ces nouvelles pratiques, qui, dans un contexte national marqué malheureusement par la prolifération des armes sur l’ensemble du territoire et leur utilisation croissante, mettent sans aucun doute en péril la sécurité nationale.

Vous citez le démantèlement d’un réseau à Marseille au mois de février 2024 par la gendarmerie nationale. Vous avez là une partie de la réponse à vos préoccupations. Les services de police et les unités de gendarmerie sont présents sur l’ensemble du spectre des trafics d’armes et déploient des savoir faire reconnus sur le terrain comme dans le cyberespace. J’ajoute bien sûr à cette mobilisation les douanes. Le constat actuel conduit toutefois à penser que le phénomène demeure contenu. D’abord, parce que certains freins technologiques limitent toujours – à moins de gros investissements – les possibilités de fabrication. Ensuite, parce que l’acquisition d’armes manufacturées reste malheureusement beaucoup plus simple pour les criminels, qu’elles soient acheminées par les filières du trafic ou issues de cambriolage de particuliers ou d’armureries. À notre dispositif opérationnel en place s’ajoute une réglementation stricte. La fabrication d’armes à feu relève de la profession d’armurier. Celui qui fabrique sans avoir ce statut tombe donc sous le coup de la loi, que l’arme soit manufacturée ou fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D. Pour aller plus loin, nous envisageons de pénaliser la fabrication, la possession et la cession par toute personne non armurier de fichiers informatiques présentant le plan de fabrication d’une arme 3D. Les discussions sont d’ailleurs engagées avec le ministère de la justice ainsi qu’avec les instances européennes dans le cadre de la prochaine directive sur l’uniformisation des infractions pénales entre États membres. La parole est à M. Pascal Savoldelli, ministre de l’intérieur. Madame la ministre, ma question porte sur les moyens de la sécurité publique en Val de Marne. La baisse de la construction de logements sociaux et l’augmentation des loyers du privé freinent l’accès aux logements des agents de police en banlieue proche de Paris.

élus, habitants et agents de police se sont réjouis du début des travaux de rénovation du commissariat au mois de septembre 2024, fruit d’une longue mobilisation. Pour autant, la question des effectifs et de la proximité reste entière.

date ? La parole est à Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Pascal Savoldelli, vous le savez, la répartition des effectifs au sein des commissariats de police tient compte de la population et des enjeux de sécurité qui sont propres à chaque territoire. le modèle spécifique d’organisation de la préfecture de police présente la particularité d’intégrer, sous l’autorité du préfet de police, l’ensemble des services de police qui œuvrent à la sécurité des habitants. Les directions ou les brigades spécialisées de la préfecture peuvent donc à tout moment intervenir sur les territoires des communes de l’agglomération parisienne, permettant ainsi de renforcer, si besoin, la présence de voie publique, y compris les unités de force mobile. Il s’agit de rechercher évidemment une plus grande efficacité. Ce modèle d’organisation,

ont fait l’objet d’importants travaux d’investissement et d’exploitation, notamment dans le cadre des jeux Olympiques. Cependant, les projets de rénovation lourde ou de restructuration, comme vous l’avez noté, ne peuvent aboutir dans un temps court. Ils font l’objet aujourd’hui de négociations pour définir les priorités. Il n’en reste pas moins que les efforts conduits

de porter un couteau traditionnel pourrait désormais entraîner une amende de 500 euros et une mention au casier judiciaire s’est propagée en Aveyron, suscitant incompréhension, interrogation et inquiétude. En effet, le couteau pliant de poche, le Laguiole par exemple, est un objet patrimonial vivant, issu de savoir faire traditionnels et artisanaux, de fabrication locale. C’est aussi un ustensile profondément enraciné dans notre culture territoriale. Le couteau est un outil usuel du quotidien que chacun utilise à table, mais aussi comme un instrument utilitaire. En milieu rural, avoir son couteau dans la poche est souvent plus utile qu’avoir un portable. dans les territoires ruraux, l’idée de sanctionner le port du couteau apparaît comme totalement inopportune et serait vécue comme une atteinte à la liberté et au mode de vie en ruralité. Madame la ministre, pouvez vous me confirmer que le port d’un couteau dans l’espace public n’est pas automatiquement sanctionné ? La sanction dépend du contexte, notamment si ledit couteau est porté dans les lieux où la loi interdit le port d’arme. Le critère déterminant est la légitimité du port dans un contexte spécifique. Le couteau Laguiole, qui est un couteau pliant à lame fixe, n’est donc pas considéré comme une arme par nature ; il peut être classé comme une arme par destination selon le contexte d’utilisation. La subtilité consiste donc à différencier la légitimité, au regard de la loi, du contexte pour déterminer si le port de l’objet est légal ou sanctionnable, ce qui n’est pas toujours évident. En effet, le dernier paragraphe de l’article 317 8 du code de la sécurité intérieure mentionne « le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros » en cas de remise volontaire à l’agent verbalisateur, « aux fins de transfert de propriété à l’État et de destruction éventuelle

Le couteau de poche traditionnel peut être apprécié comme un outil utilitaire de la vie rurale. La notion d’appréciation est précisément au cœur de la réglementation qui encadre le port des articles de coutellerie. Seuls les poignards et les couteaux poignards, se distinguant notamment par un tranchant sur chaque côté de la lame, sont expressément visés par le code de la sécurité intérieure et classés en catégorie D : ils ne peuvent être vendus qu’à des majeurs et dans des commerces ayant été autorisés par le préfet. Leur port et leur transport sont formellement interdits sauf motif légitime, comme le fait de se rendre à une action de chasse ou de reconstitution historique. Les autres couteaux, notamment ceux que vous citez et qui reflètent la richesse artisanale de nos régions, ne sont pas expressément classés dans cette catégorie. Toutefois – l’actualité nous le rappelle trop souvent –, ils sont susceptibles de blesser, voire de tuer, si on les détourne de leur usage. C’est en cela qu’ils peuvent être appréciés, en cas de contrôle, comme des armes blanches

Le recours à la procédure expérimentale de l’amende forfaitaire délictuelle repose sur les mêmes principes. Il s’inscrit dans le cadre de la politique pénale locale, qui s’assure du discernement des intervenants. La parole est à Mme Christine Herzog,

Face à l’augmentation de la délinquance et des violences urbaines, face à la progression du narcotrafic et à l’ensauvagement de la population, les policiers municipaux sont les premiers sur le terrain.

Opter pour des solutions judiciaires, c’est choisir un modèle plus répressif, qui changerait le rapport des policiers municipaux au public ; ce n’est pas forcément ce que souhaitent les élus.

aux préfets d’en faire un axe fort de leurs plans d’action départementaux de restauration de la sécurité du quotidien. Je n’irai pas jusqu’à parler d’interopérabilité, car bien des éléments singularisent

Les conclusions du Beauvau des polices municipales, mené par François Noël Buffet, sont attendues pour le début du mois d’avril prochain. Le renforcement des dispositifs de coordination figure parmi

années. Conscient de cet enjeu, l’ancien ministre de l’intérieur Gérald Darmanin avait décidé une offensive contre les incivilités, en promettant dès 2022 la création de soixante dix sept unités dédiées à la sécurisation des transports,

promulgué le 24 janvier 2023, ne fait aucune mention des effectifs supplémentaires affectés à ces brigades. Malgré les promesses gouvernementales, aucune brigade de sécurisation des transports en commun ne s’est, à ce jour, matérialisée au Mans,

pour minimiser leur impact sur les voyageurs, le Gouvernement a veillé à maintenir des dessertes ferroviaires aux heures de pointe du matin et du soir. Vous évoquez le rétablissement d’une liaison aérienne entre Limoges et Paris comme solution de substitution. La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a étudié en détail les différentes options qui s’offrent à nous. À cet égard, plusieurs obstacles juridiques et pratiques doivent être pris en compte. Premièrement, les obligations de service public (OSP) sur cette liaison sont aujourd’hui éteintes ; elles devraient être entièrement redéfinies pour s’adapter aux besoins spécifiques de cette période de travaux.

pourrait être mise en œuvre plus rapidement. Nous travaillons avec les acteurs concernés pour définir un programme de vols adapté et étudier les différentes formes de soutien possibles dans le respect du droit européen. le ministre des transports et ses services restent pleinement mobilisés pour accompagner les collectivités territoriales dans la recherche d’une solution. Il convient d’assurer au mieux la connectivité du territoire pendant cette période de travaux, tout en respectant le cadre juridique et budgétaire qui s’impose à nous. La parole est à M. Christian Redon Sarrazy, pour

Cette politique est d’autant plus problématique qu’elle s’accompagne d’une réduction de l’offre. En effet, le déclassement de 100 rames en parfait état en 2013 et le transfert récent de 14 rames Duplex en Espagne ont considérablement réduit notre capacité.

Comment le Gouvernement entend il garantir une politique tarifaire permettant réellement l’accès au train pour tous ? Comment comptez vous accélérer le renouvellement du parc de rames TGV et assurer que les choix stratégiques de la SNCF s’alignent sur les besoins des Français ? Enfin, n’est il pas temps de repenser le modèle de financement de notre réseau ferroviaire,

En tant qu’opérateur d’un service librement organisé, la SNCF dispose d’une autonomie de gestion pour fixer sa politique tarifaire, gérer son parc de matériel roulant et adapter son offre de transport à grande vitesse. Si les prix des services ferroviaires librement organisés ont fortement chuté du fait de la crise sanitaire, ils ont fait l’objet d’un rattrapage de l’indice des prix à la consommation en 2023. Pour l’année 2025, en revanche, les prix des cartes Avantage, de la carte Liberté ainsi que des abonnements Max Jeune et Senior seront gelés.

SNCF Voyageurs a fortement développé l’offre Ouigo, qui permet de proposer des trajets à prix bas pour plus de soixante destinations. En 2025, plus de la moitié des billets Ouigo seront à moins de 30 euros.

le régime de la CNRACL affichait un déficit de 3,8 milliards d’euros en 2024, mais l’augmentation des cotisations employeur est elle, pour le Gouvernement, le seul moyen d’y faire face dans la durée

Sans ces prélèvements répétés, la CNRACL disposerait de réserves suffisantes pour les dix prochaines années, à taux de cotisations constants. Le Gouvernement entend il ouvrir un dialogue de fond

Afin d’apporter une première réponse à cette situation d’urgence, le Gouvernement a décidé, par décret en date du 30 janvier 2025, d’augmenter de trois points par an pendant quatre ans, de 2025 à 2028, le taux de cotisation des employeurs.

À titre de comparaison, l’emprise foncière de la ligne entre Tours et Bordeaux représentait 13 hectares par kilomètre de voie ferrée construite, d’après un calcul de grillage à grillage, comme le prévoit la loi portant lutte Un décret d’application de cette loi qualifie en effet d’artificialisées « les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée Une modification non justifiée du mode de calcul a ainsi permis de diviser par quatre la surface artificialisée entre deux projets comparables. C’est là une entorse majeure à la loi Climat et Résilience, dont l’objectif est d’atteindre le zéro artificialisation nette des sols d’ici à 2050. Pour que la loi soit respectée, le terre plein de sécurité autour des rails soit aurait dû être compté comme surface artificialisée pour les deux projets, soit n’aurait dû l’être pour aucun des deux. deux. Madame la ministre, je demande au Gouvernement de revoir le mode de calcul de la surface artificialisée, conformément à la loi Climat et Résilience, et de réévaluer l’impact environnemental du GPSO en utilisant la méthode de décompte appliquée pour la ligne Tours Bordeaux. La parole est à Mme la ministre.

La méthode actuelle de calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers repose sur la comptabilisation des espaces effectivement urbanisés.

J’en viens au détail de ce calcul. Le décompte de 740 hectares pour le GPSO correspond à une simple estimation du programme de travaux en Nouvelle Aquitaine, pour 491 hectares, et en Occitanie, pour 249 hectares. Cette estimation inclut la plateforme ferroviaire, les raccordements, les voies d’accès et les ouvrages annexes. À l’inverse, les surfaces végétalisées des abords de l’infrastructure, qui peuvent constituer des espaces naturels, ne sont pas comptabilisées, dès lors que nous restons en mode de comptabilisation dit des Enaf. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, de revoir le mode de calcul retenu pour ce projet. S’agissant plus largement de notre capacité à respecter le forfait de 12 500 hectares,

afin de s’assurer du respect des objectifs de la loi Climat et Résilience.

cette dégradation devrait se poursuivre, puisque la SNCF vient de nous annoncer de nouvelles suppressions de trains, comme c’est le cas chaque mois désormais. Pourtant classée par l’État comme axe d’intérêt national,

Aux difficultés techniques dues au sous investissement chronique s’ajoute une pénurie de personnel. Le nombre d’agents de la SNCF est en constante diminution, tandis que les moyens nécessaires pour compenser les défaillances techniques et les pannes de locomotives ne cessent d’augmenter.

Pour autant, quelles mesures concrètes le Gouvernement entend il prendre pour assurer un niveau de service acceptable, d’ici à la modernisation effective de la ligne Polt et à la livraison des rames Oxygène, en 2027 ?

que l’État, en tant qu’autorité organisatrice, est pleinement mobilisé pour améliorer durablement la qualité de service sur la ligne Paris Orléans Limoges Toulouse. L’État a engagé un programme d’investissement sans précédent de 1,9 milliard d’euros sur la période 2018 2027 pour la régénération et la modernisation de la ligne. Ces travaux, qui avancent conformément au calendrier prévu, permettront d’améliorer significativement la régularité et les temps de parcours. Par ailleurs, nous avons investi 400 millions d’euros dans l’acquisition de vingt huit nouvelles rames Oxygène qui remplaceront progressivement le matériel actuel à partir du printemps 2027. Aussi, concernant les perturbations actuelles, la SNCF a lancé un plan d’action qui a déjà permis d’augmenter la régularité de près de 8 points par rapport à 2023, avec 83 % des trains arrivant à l’heure.

compositions renforcées pour limiter la gêne pour les voyageurs. Je précise également que le schéma directeur prévoit, à partir du mois de décembre 2027, le passage à

des habitants des territoires ruraux qui supporteront mal de voir des camions remplis de bois issu de leurs forêts partir alimenter des industries à des centaines de kilomètres, pendant que leur sera dénié le droit d’utiliser eux mêmes la biomasse pour se chauffer. Madame la ministre, le Gouvernement va t il donc persister dans cette stratégie qui privilégie la décarbonation des industries

et des tensions apparaîtront dès 2030, selon les différents scénarios de la planification écologique. Pour garantir notre souveraineté énergétique et préserver cette ressource précieuse, nous devons prioriser les usages les plus efficaces. La troisième stratégie nationale bas carbone (SNBC) titre que la chaleur haute température pour l’industrie et les réseaux de chaleur est prioritaire, tandis que le chauffage résidentiel doit être développé de manière raisonnée. Nous aurons aussi un fort besoin de biomasse pour la construction, qui devra se décarboner massivement. C’est pourquoi nous avons décidé de réduire progressivement et de façon modérée, à hauteur de 30 %, les aides MaPrimeRénov’ pour les équipements de chauffage au bois.

une aide financière pour l’accès à ce mode d’énergie. Nous continuons de soutenir la filière bois énergie et encourageons les solutions de substitution comme les pompes à chaleur, la géothermie et le solaire thermique. Nous devons agir de manière responsable et stratégique pour assurer une transition énergétique durable et équitable pour tous,

J’ai été alerté sur la nécessité de clarifier la réglementation liée à l’article R. 412 127 du code des communes dans sa version en vigueur depuis le 16 mai 1981.

Toutefois, l’interprétation de la réglementation peut laisser penser que la présence de ces agents serait uniquement obligatoire dans les classes maternelles accueillant des enfants de 3 à 5 ans. ans. Dans les milieux ruraux où les effectifs sont limités, les classes maternelles sont souvent remplacées par des classes enfantines, ce qui leur permet d’accueillir un panel plus large d’enfants âgés de 4 à 7 ans. C’est la raison pour laquelle il convient d’éclaircir la question du caractère obligatoire de la présence d’un Atsem dans les classes enfantines. Ainsi, madame la ministre, pourriez vous préciser l’interprétation de la réglementation en vigueur afin d’apporter une réponse aux acteurs engagés pour l’éducation de nos enfants dans les milieux ruraux ? La parole est à Mme la ministre.

Ils sont notamment « chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants », d’après l’article 2 du décret n° 92 850 du 28 août 1992 Par ailleurs, l’article R. 412 127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’une personne occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines La classe enfantine étant le degré intermédiaire entre l’école maternelle et l’école primaire, l’obligation de présence d’Atsem s’étend donc à ce type de classe. Je vous rappelle en tout état de cause que le recrutement et l’affectation des Atsem relèvent de la seule compétence du maire,

La séance est suspendue.